L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre

aux ordonnances prises sur le fondement de la loi d'habilitation du 15 septembre 2017, à travers le vote définitif du présent projet de loi de ratification. Ce texte constitue une réforme du droit du droit du travail sans précédent depuis trente ans, car il donne une place centrale à la négociation d'entreprise, il modernise la représentation du personnel dans l'entreprise, il sécurise les procédures de licenciement et il adapte les règles de prévention des risques professionnels. Dès l'examen du projet de loi d'habilitation, cet été, nous avions exprimé notre satisfaction de constater que le Gouvernement reprenait à son compte la plupart des des thèmes sur lesquels la majorité sénatoriale s'était mobilisée depuis 2014, comme l'assouplissement des règles du mandatement syndical, la simplification des accords de flexisécurité, la rationalisation des institutions représentatives du personnel, ou encore la remise à plat du compte pénibilité. La persévérance du Sénat porte aujourd'hui ses fruits, et confirme la pertinence de notre diagnostic et des propositions que nous formulions alors pour moderniser notre droit du travail. À l'issue de nombreuses rencontres bilatérales avec les partenaires sociaux représentatifs entre juin et septembre dernier, le Gouvernement a élaboré cinq ordonnances qui respectent globalement le cadre fixé par le Parlement dans la loi d'habilitation. En dépit de ce satisfecit général, près de 80 amendements ont été adoptés au Sénat pour enrichir le présent projet de loi, avec quatre objectifs la simplification des normes, le renforcement de la compétitivité de l'économie, la prise en compte des spécificités des petites entreprises et la protection des droits fondamentaux des salariés. Plusieurs apports décisifs du Sénat ont été conservés par la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 31 janvier dernier, et je voudrais à cette occasion saluer le rapporteur de l'Assemblée nationale, Laurent Pietraszewski, pour son écoute et son implication, ainsi que Mme la ministre et ses services pour leur disponibilité et leur engagement. Tout d'abord, la commission mixte paritaire a confirmé l'obligation de créer une commission des marchés chargée de fixer des critères objectifs pour choisir les prestataires des comités sociaux et économiques de grande taille. Les règles applicables à la nouvelle instance unique de représentation du personnel en matière de transparence financière ne pouvaient pas être moins rigoureuses que celles en vigueur depuis quatre ans dans les comités d'entreprise. Comme le souhaitait le Sénat, tous les CSE dépassant certains seuils devront être dotés d'une telle commission, sans pouvoir s'en dispenser par accord collectif. paritaire a accepté de rendre obligatoire la formation de tous les membres du CSE aux problématiques de santé et de sécurité au travail, alors que la deuxième ordonnance la réservait aux seuls membres de la commission dédiée. Cette mesure devrait être de nature à rassurer les personnes inquiétées par le transfert, pourtant à droit constant, des missions du comité Par ailleurs, la commission mixte paritaire n'a pas remis en cause la règle introduite au Sénat selon laquelle toute fraude rendait caduque l'utilisation d'un périmètre national pour apprécier, au sein d'un groupe, la cause économique d'un licenciement. paritaire a approuvé la suppression des instances de dialogue social dans les réseaux de franchise, introduite au Sénat sur l'initiative du groupe du RDSE et de plusieurs membres de la délégation aux entreprises. paritaire a maintenu les dispositions introduites au Sénat qui répondaient à des situations d'urgence. Je pense notamment aux règles relatives au développement de la mobilité européenne des apprentis, qui devaient être clarifiées rapidement pour que les apprentis puissent bénéficier dès cette année des fonds européens du programme Erasmus Pro. Je pense surtout à l'assouplissement, à titre exceptionnel et temporaire, de plusieurs règles relatives à la rupture du contrat de travail dans les collectivités ultramarines de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui ont été touchées par l'ouragan Irma, le 6 septembre dernier. Mes échanges avec le rapporteur de l'Assemblée nationale ont également permis d'élaborer des rédactions de compromis entre nos deux assemblées sur plusieurs sujets. Nous avons tout d'abord trouvé un terrain d'entente concernant la dénomination du nouvel accord de flexisécurité unique. Nous avions opté au Sénat pour le nom d'« accord de performance sociale et économique », mais nous avons finalement retenu en commission mixte paritaire celui d'« accord de performance collective afin de mettre l'accent sur la place éminente qu'il a vocation à occuper dans l'entreprise, comme c'est déjà le cas en Allemagne. S'agissant de l'interdiction d'exercer plus de trois mandats successifs de représentant du personnel, le Sénat s'était opposé à la possibilité de contourner cette règle par accord collectif dans les entreprises employant plus de 50 salariés. a rétabli cette dérogation, mais l'a circonscrite aux entreprises employant entre 50 et 300 salariés, compte tenu de la difficulté pour certaines d'entre elles de trouver de nouveaux candidats pour occuper des fonctions de représentant du personnel. Soucieux de ne pas laisser les salariés et les employeurs dans une longue période d'insécurité juridique en cas de recours en nullité à l'encontre d'un accord d'entreprise, le Sénat avait fixé au juge un délai de trois mois

Tout d'abord, la commission a rétabli la généralisation des accords majoritaires dès le 1 mai 2018, au lieu du 1 septembre 2019, comme le prévoyait la loi Travail. Le Sénat n'a de cesse de mettre en garde le Gouvernement sur le fait que cette mesure pourrait entraîner une forte diminution des accords d'entreprise, car les employeurs pourraient avoir de grandes difficultés à négocier avec des syndicats signataires réunissant au moins la moitié des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs lors des dernières élections professionnelles. Le Sénat ne s'oppose pas au principe des accords majoritaires, mais il est dubitatif quant au calendrier de leur mise en oeuvre. Je forme donc le voeu que cette mesure ne freine pas la conclusion d'accords d'entreprise, car nous partageons tous le même objectif, celui de renforcer la vitalité du dialogue social. La commission mixte paritaire a ensuite rétabli les observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Ces structures avaient été supprimées au Sénat, car aucune disposition de la loi d'habilitation n'autorisait leur création par ordonnance. Toutefois, la commission les maintenir pour faciliter le suivi des dispositions des ordonnances en faisant remonter au niveau national les éventuelles difficultés rencontrées par les employeurs et les salariés. Je rappelle à cette occasion que, si le Gouvernement doit respecter scrupuleusement le cadre fixé par la loi d'habilitation lorsqu'il rédige une ordonnance, la Constitution n'interdit pas, lors de l'examen du projet de loi de ratification, l'adoption d'amendements portant sur des dispositions non prévues par la loi d'habilitation, mais qui ont un lien, même indirect, avec son objet. Avant de conclure, je souhaiterais souligner que notre vote aujourd'hui ne mettra pas un point final à cette réforme par ordonnances du code du travail. Compte tenu de la rapidité de leur rédaction et de leur portée, il sera en effet nécessaire de leur apporter quelques corrections dans les mois et années à venir, à l'aune des observations du comité d'évaluation mis en place en novembre 2017. Le Parlement a joué pleinement son rôle dans cette réforme, en précisant le champ de l'habilitation et en modifiant les dispositions issues des ordonnances, y compris celles de la sixième, en date du 20 décembre dernier. Le succès de la réforme se mesure d'ores et déjà à l'enthousiasme que manifestent les investisseurs étrangers pour notre pays depuis son annonce. Il ne sera toutefois durable que si les partenaires sociaux s'emparent résolument des nouvelles responsabilités que leur confie la loi et si les services déconcentrés du ministère du travail accompagnent les entreprises et les salariés. À la lumière de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. La parole

monsieur le président de la commission des affaires sociales et rapporteur, cher Alain Milon, mesdames, messieurs les sénateurs, les sénateurs, « c'est là un des grands et merveilleux caractères des beaux livres que pour l'auteur ils pourraient s'appeler " Conclusions " et pour le lecteur " Incitations je crois que cette phrase de Marcel Proust synthétise d'une certaine manière l'esprit de cette lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de ratification des ordonnances pour le renforcement du dialogue social. cette séance constitue l'aboutissement du travail législatif intense que nous avons entrepris ensemble depuis juillet dernier, en faveur de plus de liberté et de plus de protections grâce à un dialogue social renforcé et décentralisé au plus près du terrain.

paritaire témoigne d'une ambition commune et partagée pour une réforme du code du travail d'une ampleur inégalée depuis une trentaine d'années. Cela tient à votre connaissance à la fois politique et technique de ce sujet passionnant, mais quelquefois complexe, sur lequel nombre d'entre vous ont travaillé lors du précédent quinquennat, que ce soit dans cet hémicycle ou dans vos circonscriptions, d'autres s'y étant plongés pleinement au cours des derniers mois. Je pense en particulier au président et rapporteur Alain Milon, dont je salue l'esprit constructif et la qualité de l'écoute et du dialogue tout au long de nos travaux. Je tiens aussi à remercier les présidents et présidentes de séance, car ils ont veillé à ce que nos débats se déroulent dans un climat serein, propice au travail de fond. Je remercie également les services de la séance et les huissiers, qui ont organisé la discussion des amendements avec une efficience remarquable, notamment lors des scrutins publics, qui requièrent une technique particulière. Enfin, je tiens enfin à saluer les administrateurs de la commission des affaires sociales pour leur disponibilité sans faille et leur vigilance précieuse quant à la qualité légistique des textes que nous façonnons ensemble. Grâce à vous tous, la discussion parlementaire, menée en parallèle d'une intense concertation avec les partenaires sociaux, a abouti au large accord trouvé en commission mixte paritaire le 31 janvier dernier. À quelques exceptions près- je pense notamment aux observatoires départementaux et au calendrier de généralisation des accords majoritaires -, cet accord reprend, comme vous l'avez relevé, monsieur le rapporteur, les évolutions introduites au Sénat en première lecture. J'en citerai quelques-unes : l'obligation d'une commission des marchés au sein du comité social et économique ; la formation obligatoire de l'ensemble des membres du CSE aux problématiques de santé et de sécurité au travail, qui me paraît être une avancée importante ou encore les dispositions visant à sécuriser juridiquement la mobilité internationale des apprentis, que nous avons élaborées un peu dans l'urgence, mais avec une vision de long terme partagée. Cet accord en commission mixte paritaire a, en outre, permis de trouver une position commune sur la limitation dans le temps de la succession des mandats des élus syndicaux. Ainsi, cet accord témoigne de la convergence renouvelée du Sénat et de l'Assemblée nationale quant à l'urgence, si j'ose dire, d'agir sur le long terme, après la succession d'échecs ou de semi-échecs collectifs à changer le regard sur l'entreprise, le but étant d'instaurer un climat de confiance indispensable au dialogue social et à la création d'emploi. C'est pourquoi l'accord en commission mixte paritaire entérine, tout en le précisant, le cadre que nous avions élaboré en ce sens, les ordonnances, comme nous nous y étions engagés devant la représentation nationale et nos concitoyens. Ce cadre juridique, vous le savez, c'est celui qui instaure depuis la parution des ordonnances les conditions d'un dialogue social structuré, lisible et décentralisé, au plus près du terrain, c'est-à-dire au plus près des entreprises et des salariés, offrant plus d'agilité et de sécurité tant aux employeurs qu'aux salariés et à leurs représentants. Tous seront des acteurs responsabilisés, davantage formés et mieux armés pour négocier, dialoguer et envisager l'avenir avec confiance. J'ai un seul regret- vous ne serez pas surpris de mes propos, puisque je l'avais déjà clairement exprimé en première lecture -, je déplore que le dispositif mis en place en 2016 pour favoriser le dialogue social dans le secteur de la franchise n'ait pu être rétabli en

Nous devrons donc travailler avec la profession à trouver une solution satisfaisante, alors que des négociations avaient été engagées par les partenaires sociaux du secteur. Enfin, cet accord en commission mixte paritaire est fondamental, car il entérine un autre engagement, important, du Gouvernement : celui d'autoriser l'assouplissement, à titre exceptionnel et temporaire, de plusieurs règles relatives à la rupture du contrat de travail dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dévastées par l'ouragan Irma. Cet engagement, que j'avais annoncé lors de mon déplacement dans les Antilles en décembre dernier, ne pouvait évidemment pas figurer dans la loi d'habilitation. Nous avons alors saisi le premier véhicule législatif pour y introduire cet amendement.

Les acteurs ont donc, grâce à la méthode retenue, d'ores et déjà la possibilité de saisir les opportunités offertes par cette réforme d'une ampleur inédite. En effet, les ordonnances, les décrets et, dans quelques heures, la loi de ratification formeront un ensemble législatif et réglementaire complet. a aussi des innovations. Je pense notamment au choix audacieux que nous avons fait ensemble de créer un droit au télétravail, particulièrement apprécié en zone rurale

Enfin, il me semble que le sens profond du vote auquel vous allez procéder dans quelques instants est celui d'un encouragement appuyé aux acteurs. C'est un signal fort envoyé à nos concitoyens, car vous leur témoignez solennellement votre confiance en leur capacité à trouver, par un dialogue social de qualité, la façon de faire converger performance économique et progrès social. Quelle est la plus belle preuve de confiance, si ce n'est la responsabilisation ? Il s'agit de donner à ceux en qui nous croyons les moyens de parvenir aux solutions adaptées à leurs attentes pour qu'ils tirent le meilleur des mutations économiques, sociales et technologiques

Vous leur demandez de rendre pleinement effectif le premier volet de la transformation profonde de notre modèle social. En leur faisant confiance, vous les rendez responsables. C'est ce que nous observerons attentivement mission que nous avons d'ores et déjà confiée à Sandrine Cazes, de l'OCDE, Jean-François Pilliard, qui est issu du monde patronal, et Marcel Grignard, qui vient du monde syndical, pour qu'ils évaluent avec les partenaires sociaux, de façon transparente et efficace, les effets de cette loi.

Ils nous disent que les discriminations dans le monde du travail ne sont plus supportables. En somme, ils nous disent que la promesse républicaine d'émancipation individuelle et collective est grippée ou insuffisante. D'où l'impérieuse nécessité de poursuivre la transformation en profondeur de notre modèle social, celle que nous avons justement engagée ensemble avec les ordonnances. Aussi, pour que la croissance soit pleinement inclusive que le travail puisse être facteur de réalisation pour le plus grand nombre, il nous faut doter nos compatriotes, à travers les compétences, non seulement d'une protection plus efficace contre le chômage et la précarité, mais aussi d'un véritable levier pour leur permettre choisir leur avenir professionnel. est le sens du plan d'investissement dans les compétences, doté de 15 milliards d'euros. Cet investissement massif et sans précédent sera accompagné des transformations tout tout aussi ambitieuses de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage, que nous avons soumises à la concertation. Elles constitueront, vous le savez,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a achevé le processus de ratification des ordonnances choisi par le Gouvernement. Nous continuerons à dénoncer cette procédure qui prive la représentation parlementaire de nombreux moyens de contestation et de proposition. Pour ne prendre qu'un exemple, votre gouvernement a réussi à faire adopter, le 24 janvier, une sixième ordonnance, déposée sous forme d'amendement en séance, sans que ni la commission des affaires sociales du Sénat, ni l'Assemblée nationale, ni encore moins les syndicats de salariés, aient eu leur mot à dire.

par la commission mixte paritaire. Là encore, on est loin de la simple correction d'une erreur matérielle ou d'un amendement de clarification. Il s'agit Il s'agit d'un recul grave pour la protection de milliers de salariés, et notamment de cadres. Je rappelle qu'actuellement l'accord du salarié est obligatoire et que, s'il refuse de signer une convention individuelle de forfait, l'employeur ne peut ni appliquer d'office le forfait ni sanctionner l'intéressé. Il doit soit renoncer à son projet, soit engager une procédure de licenciement, selon la décision de la Cour de cassation du 30 mai 2007. Tout cela vole en

Cette nouvelle norme entravera encore plus les moyens d'action des salariés sur un sujet fondamental : la remise en cause d'avantages garantis jusqu'à présent par les branches. La commission mixte paritaire a également tranché en faveur de l'extension de la rupture conventionnelle collective aux entreprises dépourvues de comité social et économique, alors que la version du Gouvernement elle-même n'allait pas jusque-là. De plus, la limitation à trois mandats successifs pour les représentants des salariés a encore été aggravée. Alors que le Gouvernement souhaitait offrir la possibilité

Comment ne pas interpréter ce nouveau recul comme une traduction supplémentaire de la volonté d'affaiblir la représentation des salariés, en la privant de ses éléments les mieux formés et les plus aguerris tout en plongeant les nouveaux venus dans des instances plus complexes, avec moins d'heures de représentation et de moyens d'action

Vos beaux discours sur la modernisation du dialogue social s'envolent donc lorsqu'il s'agit de préserver les intérêts des grands groupes, lesquels pourront, de fait, mettre en oeuvre la rupture conventionnelle collective quand bon leur semble. C'est vrai, vous prétendez éviter le « traumatisme du licenciement », mais les salariés, grâce à vous, ou plutôt à cause de vous, pourront se retrouver à la rue sans accompagnement, en contrat de sécurisation professionnelle et sans priorité de réembauche. Voilà le changement Je pense ainsi à l'entreprise Téléperformance, qui envisage de se débarrasser de 240 salariés une rupture conventionnelle collective avec, pour seul accompagnement, mois de salaire net pour tous et une prime d'incitation de 2 000 euros à 10 000 euros suivant l'ancienneté ; bref, un dispositif évidemment moins lourd et moins cher qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, mais qui a vocation à se généraliser, avec à chaque fois la même finalité- nous ne pouvons que le déplorer -, la suppression d'emplois pour renforcer la profitabilité de l'actionnariat. La vérité, c'est que toutes ces mesures régressives que j'ai énoncées réduisent encore plus les protections des salariés et sécurisent abusivement, parfois, la situation des employeurs

plus lisible, à la fois protecteur pour les salariés et garant de l'efficacité économique. Ce n'est pas le chemin que vous avez choisi, vous avez préféré vous appuyer sur le libéralisme assumé de la majorité sénatoriale pour vous éloigner encore plus des déclarations d'intention que vous aviez faites, à l'origine, à l'attention des syndicats de salariés. À l'arrivée, votre projet de loi choisit clairement son camp ; nous nous y opposerons frontalement par notre vote

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le 24 janvier dernier, le Sénat adoptait le texte du projet de loi ratifiant les ordonnances pour le renforcement du dialogue social, enrichissant ce texte au travers de plus de 70 amendements.

je tiens ici à saluer le travail de l'ensemble de nos collègues parlementaires, grâce auxquels ce texte a pu aboutir. Si la réforme du code du travail était attendue, elle suscitait toutefois des craintes. Les ordonnances ainsi ratifiées apportent des garanties tant aux employeurs qu'aux salariés, pour lesquels il était essentiel d'intégrer des mesures d'accompagnement et de protection. La version issue de nos travaux a su trouver un juste équilibre entre le respect du cadre fixé par la loi d'habilitation et son adaptabilité aux exigences actuelles de notre économie et de ses acteurs, nos entreprises. Si le champ des habilitations devait être respecté, il était en effet impératif d'intégrer des dispositions nouvelles pour faire face à des situations particulières.

D'autres mesures adoptées par la commission mixte paritaire méritent d'être soulignées. L'appellation finale retenue pour l'accord de performance en fait partie. Ce nouvel accord de flexisécurité, qui harmonise les accords précédents, avait été renommé « accord de performance sociale et économique » par la Haute Assemblée. La commission mixte paritaire, quant à elle, a retenu l'appellation d'« accord de performance collective ». Ce choix nous satisfait en grande partie, car il préserve la notion de performance, à laquelle le Sénat était attaché. Au-delà du terme choisi, il convient de rappeler qu'une étape importante est franchie, car ce nouvel accord permettra aux entreprises de réagir plus rapidement et avec plus de souplesse aux fluctuations et aux exigences économiques. Un autre sujet sur lequel la commission mixte paritaire a dû trouver un accord, après de nombreuses discussions, porte sur la limitation dans le temps des mandats des élus syndicaux. Nous avions fait le choix de supprimer la possibilité de déroger à cette limitation. L'impératif de renouvellement des instances représentatives du personnel était, à nos yeux,

La commission mixte paritaire a cependant adopté la possibilité de déroger à cette limitation, cela a été rappelé, pour les entreprises dont les effectifs sont compris entre 50 et 300 salariés. Nous espérons que cette disposition ne freinera pas le nécessaire renouvellement des élus syndicaux En définitive, ces ordonnances, telles qu'elles résultent de ces deux mois de débat, actent le début d'une réforme attendue par nos entreprises, pour lesquelles la consécration du principe de subsidiarité, par défaut de l'accord d'entreprise ou encore l'application d'un barème impératif de dommages et intérêts sont autant de gages de sécurité. Cette refonte de notre architecture conventionnelle profitera également aux salariés, grâce au renforcement du rôle des branches, dont les accords primeront dans treize domaines, et à l'instauration de la nouvelle règle majoritaire, qui permettra de sécuriser les relations entre salariés et employeurs. Mes chers collègues, ces ordonnances marquent le début d'une réforme plus générale de notre modèle social. Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la discussion du texte en première lecture, il sera nécessaire de repenser des mesures sécurisant les parcours professionnels. Ce sera l'objet des réformes à venir, celle de la formation professionnelle et de l'apprentissage, dont les orientations viennent d'être présentées par le Gouvernement. Gardons toutefois à l'esprit que notre volonté est de poursuivre la simplification des textes pour leur meilleure application. En parallèle, je l'avais abordé préalablement, je pense que la médecine du travail devrait faire l'objet d'une attention toute particulière. Elle doit retrouver tout son sens du point de vue de la prévention et de la protection des salariés.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, sociales, mes chers collègues, voici donc la dernière étape du parcours des ordonnances modifiant le code du travail, et le résultat, confirmant ce que nous redoutions, est triste, régressif, attentatoire aux droits historiques conquis par les salariés. Ni révolutionnaire ni moderne, mais bien rétrograde ... Vu la finalité recherchée, le résultat ne pouvait qu'être nocif, et nous aurons, hélas, à en déplorer les effets délétères. Il sera générateur de précarité pour les travailleurs et tout à fait conforme à l'objectif annoncé : licencier plus facilement pour embaucher plus- un slogan en forme d'incantation repris et répété à l'envi, ce qui ne suffit pas à en faire une vérité, bien au contraire. Oh, les mots, pourtant, chantent dans l'exposé des motifs ! Ils prétendent à une double volonté : l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises et le renforcement de la sécurité des salariés. Or seule la première ambition trouve ici, largement, satisfaction.

La procédure imposée, celle des ordonnances, plombe un peu le débat. Les ordonnances sont appliquées depuis septembre après la seule discussion sur la proposition d'habilitation. Nulle urgence n'exigeait que l'on procédât ainsi. aucune urgence en effet, puisque la loi El Khomri, à peine portée sur les fonts baptismaux, se trouve excommuniée et remplacée par un texte dont on clame à tort qu'il la compléterait et s'inscrirait dans son droit fil. Il n'en est malheureusement rien ; il s'agit bien d'une rupture de logique, d'un renversement des valeurs exprimées dans le projet du précédent gouvernement. Ces ordonnances constituent, hélas, une construction cohérente avec vos objectifs, avec, en même temps, une forme d'angélisme mystificateur, qui s'appuie sur un postulat que nous aimerions vrai, mais qui est loin de l'être : la confiance présiderait naturellement, selon vous, à toute négociation. Or une négociation exige plus que de la confiance ; elle nécessite, pour être fructueuse et mobilisatrice, un véritable équilibre dans le rapport de forces, ce que vous détruisez avec une Dans la plupart des entreprises, notamment dans les TPE et PME, l'atmosphère peut être chaleureuse et le désir de développement partagé par l'ensemble du personnel ; pour autant, considérer que les négociations sur des sujets aussi essentiels que les conditions de travail, d'horaires, de rémunération et de licenciement, qui engagent la vie des familles, puissent ne reposer que sur une certaine confiance réciproque, quand les intérêts sont divergents, relève au minimum d'un certain aveuglement. Licencier sans trop de difficultés et réduire le coût du travail, tous les outils figurent dans la panoplie que vous avez confectionnée, madame la ministre, avec l'accord de la majorité sénatoriale. les accords d'entreprise n'impliquent plus la présence de délégués syndicaux ni de salariés mandatés. Or ces négociations totalement déséquilibrées, en raison du statut d'autorité de l'employeur de la situation de subordination des salariés, peuvent porter gravement atteinte aux revenus comme aux conditions de travail pour aboutir, dans certains cas, à des accords plus contraints que négociés. Que dire des accords de performance collective, dont on vient de se louer ? La majorité a voulu cette appellation plutôt que celle d'« accord de compétitivité ». Il ne s'agit pas seulement d'une coquetterie sémantique la compétitivité se mesure par comparaison avec les entreprises concurrentes. La performance, elle, peut relever d'une décision totalement arbitraire, tant dans ses fondements que dans ses objectifs.

d'un tel accord adopté par un référendum à la main du patron entraîne un licenciement mécaniquement réputé « pour cause réelle et sérieuse ». Alors, l'emploi peut facilement devenir la variable d'ajustement de la gestion de l'entreprise. Vous prétendez organiser le dialogue social. En réalité, ce projet étend, organise, officialise, légitime le monologue social, à telle enseigne, d'ailleurs, qu'une proposition pertinente fixant à 12 ans plutôt qu'à 3 mandats la durée maximale d'exercice des délégués du personnel a été rejetée par la majorité, alors que la durée de ces mandats varie de 2 ans à 4 ans. En 6 ans, les délégués n'auront pas trop le temps d'acquérir les connaissances, l'expérience et le savoir-faire indispensables à la pratique de la négociation et de la médiation

Si le licenciement pour cause réelle et sérieuse est impossible, malgré la facilité qu'il y a à y recourir, il reste la possibilité, sans trop bourse délier, de s'autoriser des licenciements qualifiés d'abusifs par le tribunal de prud'hommes, puisque le plafonnement des dommages et intérêts le risque financier pour l'employeur et prive le salarié d'une juste réparation du préjudice subi. Nous avons eu l'occasion de dénoncer les atteintes portées aux moyens accordés aux salariés pour agir sur la prévention des handicaps et des maladies engendrés par certains métiers exposés, alors que les conditions de travail, la pénibilité et la précarité sont à l'origine de la plus grande injustice qui soit : celle de la longévité. En effet, les pauvres vivent en moyenne 13 ans de moins que les riches ! Pourtant, vous supprimez- pardon, vous « fusionnez -les CHSCT, qui perdront leur vocation unique et efficace de prévention et de détection des conditions de travail génératrices de troubles et de pathologies graves. Quatre domaines de travaux pénibles ont été retirés de la liste ; triste décision, qui ne contribuera pas à atténuer les inégalités insupportables que je viens d'évoquer.

parce que, ainsi, la clarté est faite sur la disparition de l'ambition de prévention au profit de la seule réparation. que dire de la méthode utilisée pour faire adopter une sixième ordonnance, sans loi d'habilitation, sans grand débat, juste au travers d'un amendement insérant un article additionnel pour faire approuver, contrairement à vos affirmations, des modifications substantielles ? Il est tout de même inouï de constater que l'Assemblée nationale n'aura jamais eu à en débattre voilà donc presque au terme du voyage effectué par les ordonnances ; permettez-moi d'en tirer quelques enseignements. Dans une France qui renoue avec le dynamisme économique grâce aux efforts consentis au cours des années précédentes, il y avait sûrement plus urgent que de casser ce qui protégeait les travailleurs français- les plus productifs au monde -, en précarisant leur situation. Les différentes mesures de ce projet de loi conduiront, au moins dans un premier temps, à des vagues de licenciements. Nous aurions dû prendre de temps de méditer les conséquences des dérégulations en Allemagne : des à un euro, des temps très partiels non voulus, des emplois précaires pour 7 7 600 000 personnes ... Est-ce donc le modèle que nous souhaitons nous donner ? Il y a fort à parier que les mesures fiscales et la dérégulation du code du travail déboucheront sur des inégalités plus grandes, ce que relève Patrick Artus, responsable chez Natixis est loin d'être un dangereux gauchiste ... Celui-ci précise : « On observe bien aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, la succession d'évolutions que Karl Marx avait prévues. » La limite est « atteinte quand les bas salaires deviennent trop faibles, et les capitalistes se lancent dans des activités spéculatives qui font apparaître les crises financières Alors que la France renoue avec la croissance, alors que s'ouvre un horizon plus serein, il eût été juste et opportun de redistribuer les bénéfices à ceux qui ont permis que cela fût, mais votre loi ouvre la porte à la diminution du coût du travail par des accords d'entreprise forcément contagieux, tout cela au profit, pour partie, de l'augmentation des dividendes qui ont pourtant atteint, en France, des sommets mondiaux en 2017. Ainsi, c'est une occasion ratée de prendre le train du progrès social, du partage d'une même ambition, de la mobilisation de l'ensemble des acteurs qui font le dynamisme et la vitalité de notre pays. Les fruits de la croissance seront suaves pour les plus favorisés ils auront un goût amer pour les travailleurs de ce pays. Des projets de loi sur l'apprentissage, sur la formation, sur le chômage et le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises sont sur le métier espérons que l'ouvrage qui en sortira aura la beauté des mots qui les présentent, et qu'il rétablira l'équilibre entre compétitivité et avancées sociales pour les salariés. Ce n'est pas le cas

la semaine passée, l'Assemblée nationale a approuvé à une large majorité le texte issu de la commission mixte paritaire ratifiant les ordonnances sur le dialogue social. À l'occasion de ces travaux conjoints,

Cette réforme répond à une ambition largement partagée, celle de simplifier le quotidien des entreprises en modernisant les règles du droit du travail, en offrant davantage de lisibilité aux salariés comme aux employeurs, en assurant une meilleure adaptation des normes à la spécificité des entreprises, notamment des TPE et PME. Je rappelle que 4 % des entreprises de moins de 50 salariés ont un délégué syndical.

; elle facilite la mise en place d'un compte pénibilité gérable et permettant d'avoir une retraite anticipée ; elle établit un barème d'indemnités prud'homales, une mesure d'équité sur le territoire

En adoptant le texte de la commission mixte paritaire, nous achevons le processus de construction d'une nouvelle forme de dialogue social en France. D'une part, ce texte revient sur deux dispositions supprimées par la commission des affaires sociales du Sénat. Il rétablit la généralisation des accords majoritaires au 1 mai 2018 et les observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. adopte une grande partie des mesures introduites par la commission des affaires sociales du Sénat : formation de tous les délégués du CSE, maintien de l'appellation de l'accord de performance sociale et économique, de la mobilité internationale et européenne des apprentis- c'est important pour le développement de l'accès à l'emploi de nos jeunes au niveau international

dans les collectivités ultramarines de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, lourdement touchées par l'ouragan Irma. En adoptant ce texte, nous faisons évoluer positivement notre modèle social, qui conserve son socle, contribuons à renforcer notre économie. C'est une étape importante, à laquelle le groupe Les Indépendants est heureux de s'associer. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la ratification de ces ordonnances constitue un signal fort pour les entreprises de ce pays. Depuis 2000, l'emploi industriel a diminué de 25 % en France du fait du renchérissement du coût du travail et de la complexité du code du travail. feront évoluer le dialogue social dans le sens de la simplification, sans précariser les salariés. Ce texte constitue un élément important pour aller vers le plein emploi il est nécessaire, mais n'est pas suffisant. Le Gouvernement devra encore s'engager à favoriser la compétitivité des entreprises et aussi à mener à bien un autre sujet prochainement porté au débat public, celui de la formation professionnelle et de l'apprentissage, clef de voûte de l'emploi des jeunes. En attendant, le groupe Les Indépendants votera en faveur de cette loi de ratification des ordonnances sur le dialogue social. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le Président de la République déclarait, le 31 août dernier : « La réforme du marché du travail est une réforme de transformation profonde [ elle doit être assez ambitieuse et efficace pour continuer à faire baisser le chômage de masse et permettre de ne pas revenir sur ce sujet durant le quinquennat. » C'est dans cet esprit que nous arrivons aujourd'hui au terme du processus de ratification des ordonnances, qui a permis au Gouvernement de prendre des mesures

Faire preuve de pragmatisme en permettant aux entreprises de créer des emplois est une impérieuse nécessité si nous voulons combattre le chômage de masse. Notre collègue Françoise Laborde l'avait rappelé en août dernier, être au chômage implique, outre la perte de revenus, la souffrance liée à la perte d'un lien social et une atteinte à l'estime de soi. Cette loi s'inscrit dans le cadre plus large la rénovation de notre modèle social amorcée par la loi El Khomri du 8 août 2016, qui se poursuivra au travers de différents textes portant sur l'apprentissage, la formation professionnelle, l'assurance chômage, les retraites et le renforcement de la participation et de l'intéressement. Les dispositions que nous ratifions aujourd'hui répondent à la nécessité d'adapter le fonctionnement de notre économie et des entreprises aux enjeux d'une compétition internationale incontournable de vue de la compétitivité et de l'attractivité de notre pays. Ces évolutions doivent permettre de stimuler l'entrepreneuriat, l'investissement et,, le développement des entreprises qui sont- nous le savons tous -le principal moteur de la création d'emplois.

qui concerne ces ordonnances, nous nous étions déjà félicités de la volonté du Gouvernement de privilégier des mécanismes opérationnels susceptibles de trouver facilement une traduction concrète dans la négociation sociale et le fonctionnement des entreprises. Après avoir abouti, en juillet dernier, à un texte commun sur le projet de loi d'habilitation, nous arrivons aujourd'hui assez logiquement aux mêmes conclusions pour la ratification, ce qui souligne les convergences de vues entre les deux assemblées. Les désaccords, qui portaient essentiellement sur des différences d'appréciation, ne remettaient pas en cause la ligne directrice de ce texte, et la commission mixte paritaire a permis de trouver des compromis. Je tiens d'ailleurs à saluer la qualité des échanges entre nos deux chambres, qui a permis d'aboutir à un texte équilibré.

de la fusion des institutions représentatives du personnel, de la formation en matière de santé et de sécurité pour l'ensemble des membres du futur comité social et économique, de la mise en place des contrats de chantier ou d'opération, de la majoration de 25 % des indemnités de licenciement calculées sur les dix premières années d'ancienneté, de la possibilité pour le ministre du travail de refuser d'étendre un accord de branche si celui-ci n'est pas compatible avec les objectifs de la politique de l'emploi, des mesures permettant de favoriser la mobilité internationale et européenne des apprentis, des mesures exceptionnelles d'adaptation outre-mer du droit du travail, à la suite du passage de l'ouragan Irma, qui devraient offrir des réponses et un accompagnement à la hauteur des dégâts occasionnés, comme l'avait rappelé notre collègue Guillaume Arnell. nous notons avec satisfaction que la commission mixte paritaire a conservé deux amendements émanant du RDSE, le premier incluant l'aléa inhérent aux pics de pollution dans la négociation sur le télétravail, le second, défendu conjointement avec la délégation aux entreprises, supprimant la mise en place d'une instance du dialogue social dans les réseaux de franchise. Madame la ministre, vous l'aurez compris, la majorité des sénateurs du groupe du RDSE soutiendra le texte de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales et rapporteur, mes chers collègues, nous voilà parvenus au terme d'une réforme d'ampleur du dialogue social et du droit du travail, pour laquelle, n'en déplaise aux tenants du coup d'État social, le travail parlementaire a été particulièrement dense et fructueux. La réunion de la commission mixte paritaire a permis de surmonter les divergences entre les deux assemblées et d'aboutir à un texte de compromis grâce à des échanges particulièrement constructifs. Voilà une vertu du bicamérisme qu'il est toujours bon de célébrer. Il est vrai que, sur les vingt articles du projet de loi de ratification qui restaient en discussion, la convergence de vues prédominait. Seuls subsistaient quelques désaccords, liés à des questions néanmoins substantielles. Les avancées réalisées par chacune des assemblées ont été conservées. Je pense en particulier à l'abondement renforcé du compte personnel de formation dans le cadre d'un accord de préservation

ou encore à l'obligation de création d'une commission des marchés au sein du comité social et économique des grandes entreprises. Pour ce qui est des points de désaccord, la commission dans certains cas, de rétablir le texte adopté à l'Assemblée nationale, notamment s'agissant du rétablissement du calendrier d'entrée en vigueur des accords majoritaires et de la confirmation du rôle des observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social. a permis de trouver une rédaction de compromis pour le délai, fixé à six mois, dans lequel le juge devra statuer sur l'action en nullité d'un accord collectif.

pour les seules entreprises employant entre 50 et 300 salariés. Cette dérogation devra être prévue dans le protocole d'accord préélectoral. Je veux également dire un mot de l'article 14, introduit au Sénat par un amendement de notre rapporteur afin de faciliter la mobilité internationale et européenne des apprentis. Cette disposition va permettre de lever l'un des freins qui empêchent le plein essor d'Erasmus Pro. Aujourd'hui, en effet, l'apprenti envoyé à l'étranger demeure sous la responsabilité de l'employeur français. C'est pourquoi les apprentis partent généralement pour quelques semaines. Afin d'offrir aux apprentis les mêmes chances de formation qu'aux étudiants, il fallait donc aménager le contrat d'apprentissage pendant le séjour à l'étranger. C'est le sens de la disposition nouvelle, qui prévoit que, pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil sont seuls responsables des conditions d'exécution du travail. Le contrat d'apprentissage de départ est en quelque sorte suspendu sur certains Cette réforme va encourager la mobilité européenne des apprentis, sans qu'il soit besoin d'attendre la réforme de l'apprentissage, qui viendra prochainement, madame la ministre, conforter ce premier pas. Pour conclure, je dirais que, en ratifiant ces ordonnances, nous posons la première pierre de la rénovation du système social français. D'autres suivront, comme la réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle, de l'assurance chômage et des retraites. Conduites avec résolution, mais sans brutalité, ces réformes portent la marque d'une méthode de gouvernement que les Français attendaient. Bravo

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voilà parvenus à l'issue de la réforme du droit du travail promise lors de la campagne présidentielle. Les ordonnances visent deux objectifs mettre fin à l'invasion de règles qui ont progressivement étouffé nos entreprises et opérer un changement de direction pour l'économie française. Vous le savez, notre groupe propose depuis déjà plusieurs années un certain nombre de mesures pour libérer le travail. Jusqu'à présent, ces mesures n'avaient rencontré, il faut le dire, qu'un écho bien faible du côté de l'Élysée, y compris lorsque l'actuel Président de la République conseillait l'ancien L'inscription dans ce projet de loi de nombreuses dispositions que nous demandions est donc positive : barème et plafonnement des indemnités de licenciement ; choix du périmètre au niveau duquel le juge pourra apprécier les difficultés économiques d'une entreprise devant licencier fusion des instances représentatives des salariés ; réforme du mandatement syndical, essentielle pour les TPE-PME ; reconnaissance juridique des accords de flexisécurité limitation des délais de recours contre les licenciements pour motif personnel ; création d'une rupture conventionnelle collective ; suppression du contrat de génération, dont nous avions d'ailleurs prévu l'échec l'échec ; simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité, dénoncé pour sa lourdeur par l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Vous le voyez, la liste de ces mesures que nous avions tenté d'introduire dans de précédents textes Elle a été utilement complétée par le travail de notre rapporteur, dont je salue l'écoute et l'implication. Ces dispositions justifient à elles seules que nous votions ce projet de loi. Cependant, nous aurions pu aller plus loin. En effet, la route de la compétitivité des entreprises n'a pas été totalement déblayée de ses principaux obstacles. Je pense aux seuils sociaux. Rappelons que le simple passage de 49 à 50 salariés entraîne l'application de près de 34 obligations légales et fiscales supplémentaires, que l'augmentation du coût du travail et la multiplication des obligations administratives liées au dépassement des seuils empêcheraient la création de 70 000 à 140 000 emplois. Alors, pourquoi attendre ? Je pense également à la durée légale du travail et aux semelles de plomb que constituent les 35 heures. Quant à la liberté d'action des entreprises, qui devait être assurée par la primauté des accords d'entreprise, elle n'a pu totalement aboutir, puisque le Gouvernement a donné finalement la priorité aux accords de branche. ces ordonnances, bien qu'elles contiennent indéniablement de très bonnes dispositions, peuvent néanmoins créer des frustrations, chez les chefs d'entreprise, qui verront parfois leur quotidien amélioré, mais pas leur environnement transformé, chez les salariés, qui bénéficieront sans doute d'un meilleur dialogue social, mais attendent aussi un pouvoir d'achat augmenté, et chez les personnes sans emploi, qui verront certains freins au travail se lever, mais pas nécessairement des emplois à la clef. Notre pays a besoin d'un projet clair, courageux, rigoureux, pour pouvoir profiter d'une relance dont profitent déjà nos voisins. Pour cela, il faudra davantage qu'un assouplissement de la réglementation sociale et des évolutions : il faudra d'importantes réformes structurelles. Notre groupe votera ce texte, qui marque une amélioration de l'existant, mais sera attentif à ce que ces premiers pas soient suivis d'autres avancées. La discussion

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité

assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, communément dénommée « directive NIS », et une directive du 17 mai 2017 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, Ce projet s'attache également à tirer les conséquences, en droit français, d'une décision, ayant d'ailleurs valeur réglementaire, relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation

En première lecture, votre assemblée s'est efforcée, d'une part, d'assurer la conformité du projet de loi avec les directives, afin d'éviter toute sous-transposition et, d'autre part, d'améliorer la précision et l'intelligibilité du texte. L'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, conservé les apports du Sénat sur ce projet de loi, l'enrichissant d'un certain nombre d'améliorations rédactionnelles.

étendant l'incrimination relative à la tentative d'acquisition, de cession ou de détention illégale d'armes, plus particulièrement de catégorie C. Pourquoi l'Assemblée nationale avait-elle introduit ces dispositions ? Parce qu'elle avait souhaité anticiper la mise en conformité de notre droit avec un protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites

pouvaient être considérées comme plus dangereuses. L'Assemblée nationale avait rétabli le texte initial du Gouvernement, suscitant l'émoi des collectionneurs. Il nous semblait

dans le prolongement des attentats tragiques qui nous ont frappés en 2015. Le fil conducteur de ce texte révisé a été le renforcement du contrôle de la circulation et du commerce des armes à feu,

l'enregistrement des armes ; une vérification préalable à la livraison de l'identité et du titre de détention de l'acquéreur pour les ventes d'armes à distance. En pratique, vous savez que ces ventes entre particuliers devront faire l'objet d'une vérification par un professionnel préalable à la livraison pour s'assurer de l'identité de l'acquéreur et du fait qu'il n'est pas interdit de détention d'armes. qu'il n'est pas interdit de détention d'armes. Enfin, le texte permettra aux armuriers de refuser légalement de conclure certaines transactions d'armes ou de munitions qu'ils pourraient raisonnablement considérer comme suspectes, leur assurant ainsi une protection juridique qui leur fait aujourd'hui défaut. Toutes ces dispositions sont guidées par le souci de renforcer les contrôles sur la circulation et le commerce des armes, dans un but exclusif de sécurité publique. Il était nécessaire et urgent d'inscrire au plus vite ces dispositions

La CMP a trouvé un habile compromis pour concilier les intérêts des collectionneurs d'armes et les impératifs de sécurité ayant inspiré la directive de 2017. Les collectionneurs seront satisfaits du maintien du classement législatif des armes reconnues comme historiques dans la catégorie D, celle des

La principale divergence entre le Sénat et l'Assemblée nationale a porté sur l'encadrement des régimes légaux d'acquisition et de détention des armes à feu

avec attention. Ce projet de loi aura des conséquences sur l'appréhension de la cybersécurité par les acteurs économiques et appellera à un système européen de certification et à l'affirmation d'une double stratégie,

Face à l'ampleur des questions soulevées, mon collègue René Danesi et moi-même nous sommes vu confier, dans le cadre de la commission des affaires européennes, la rédaction d'un rapport sur le thème de la cybersécurité. Nous avons pour objectif de dresser un état des lieux des différents textes et pour ambition de proposer quelques pistes de travail à l'échelle européenne pour tendre vers une certification adaptée et efficace, dans un esprit pragmatique.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité regroupe trois sujets bien distincts. Il s'agit d'abord de transposer la directive 2016/1148 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, autrement dit à lutter contre la cybercriminalité au niveau européen et à garantir un niveau de sécurité élevé des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services dits essentiels. Il s'agit ensuite de transposer la directive modifiant la directive relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes en mettant en place un système de contrôle de l'acquisition et de la détention des armes à feu. Il s'agit enfin de tirer les conséquences de la décision européenne relative au fonctionnement du système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.

entre ce qui relève du domaine législatif ou du domaine réglementaire. Concernant la transposition de la directive relative à la cybersécurité, l'actualité récente a montré que tous les secteurs d'activité pouvaient être victimes d'attaques informatiques importantes, susceptibles voire de paralyser l'activité économique bien au-delà des frontières d'un État. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de ces dispositions qui visent à renforcer le niveau de cybersécurité. En effet, les cyberattaques ne cessent de s'accroître, occasionnant des dégâts très importants. Ainsi, l'attaque subie par Saint-Gobain en août 2017 aurait entraîné des pertes de 250 millions d'euros environ. Ce phénomène touche également les entreprises de taille plus réduite. Selon les estimations de la Commission européenne, l'ampleur de ces attaques informatiques est sans précédent : 80 % des entreprises européennes en seraient victimes. Dans certains États membres, la cybercriminalité représenterait 50 % des infractions constatées. Ainsi, actuellement, la cybercriminalité dispose d'un champ d'action pratiquement illimité. Face à ce constat de criminalité sans frontières, il apparaît clairement qu'aucune politique nationale ne peut à elle seule être suffisante. Pour lutter efficacement contre la cybercriminalité, une approche commune permettant une coordination est primordiale. L'obligation de respecter un socle minimal de mesures de sécurité, de contrôle et de déclaration des incidents paraît indispensable. Les dispositions prévues dans ce texte sont parfaitement adaptées à la situation actuelle. de loi donne à la France les moyens de se prémunir contre les cyberattaques en imposant aux opérateurs et aux fournisseurs de services numériques d'identifier les risques potentiels en matière de sécurité numérique, de prendre à leurs frais les décisions qui s'imposent pour les maîtriser et d'informer l'autorité nationale compétente en la matière. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, assure la défense et la sécurité des systèmes d'information, a donc par nature vocation à être au coeur du dispositif de transposition. Elle se verra ainsi attribuer de nouvelles missions.

En effet, la Haute Assemblée avait soulevé un risque d'inconstitutionnalité de cet article relatif aux obligations s'imposant aux opérateurs de services essentiels en matière de cybersécurité, tout en estimant ne pas pouvoir aller plus loin à ce stade, faute d'informations suffisantes

compromis trouvé sur le classement d'armes historiques satisfera les collectionneurs, qui étaient inquiets. La modification de l'article 16 vise à permettre que les armes historiques soient classées en catégorie D par le législateur et que les reproductions d'armes historiques et les armes neutralisées soient classées par décret en Conseil d'État. Deuxièmement, la création, souhaitée par l'Assemblée nationale, d'une infraction de tentative d'acquisition ou de cession illégale d'armes permettra à la France de se mettre en conformité avec le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu.

La loi du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif renvoyait en effet à un décret la création de cette carte de collectionneur. Enfin, je ne m'étendrai pas sur Galileo, mais je salue l'ambition de ce projet, qui permettra de mettre fin à toute dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis en matière de positionnement par satellite. La France a beaucoup investi dans ce programme, sur le plan tant financier

si certains se plaignent parfois de la surtransposition des normes européennes dans l'ordre juridique français, celles que nous transposons aujourd'hui, par le biais de cette commission mixte paritaire, sont nécessaires. Elles sont nécessaires, car elles traitent de sujets importants pour notre pays, qu'il s'agisse de la lutte contre la cybercriminalité, du renforcement du cadre de la commercialisation des armes à feu ou encore de l'exploitation des données collectées par Galileo. Elles sont nécessaires, car elles renforcent la position de pointe de la France en matière de cybersécurité. Parce que la transposition laisse souvent peu de place à l'interprétation, nous nous devions d'examiner sérieusement ces dispositions. À cet égard, je salue le travail effectué par notre rapporteur, Philippe Bonnecarrère,

des peines. L'Assemblée nationale nous a entendus et a précisé les domaines dans lesquels le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des réseaux et systèmes d'information, ce dont nous nous félicitons. Nul besoin ici de rappeler l'importance grandissante de ces sujets. Si, jadis, la cybersécurité était réservée aux techniciens, elle nous concerne aujourd'hui tous, que l'on habite à Paris, à Lyon ou bien dans les Hautes-Pyrénées- oui, on peut résider en zone blanche et être exposé à la cybercriminalité En ce sens, nous devons mener une politique ambitieuse afin de sensibiliser nos entreprises, petites et grandes, aux cyberattaques. Je rappellerai, comme l'ont déjà fait nombre de mes collègues, les estimations de la Commission européenne, alertant sur l'ampleur de ces phénomènes sans précédent 80 % des entreprises européennes seraient victimes d'attaques et, dans certains États membres, la cybercriminalité représenterait 50 % des infractions constatées. À ce titre, je tiens tout particulièrement à saluer le travail effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, laquelle, depuis 2009, apporte son expertise à nos entreprises privées comme publiques, leur permet d'assurer de manière sereine leurs missions et les accompagne lorsqu'elles sont victimes de cyberattaques. Toutefois, si je devais exprimer un regret, ce serait que notre groupe n'ait pas été entendu concernant le rôle que doit jouer l'ANSSI. Nous continuons de penser que ce texte confie de trop nombreuses prérogatives au Premier ministre. Il nous aurait semblé plus judicieux de confier ces missions à l'ANSSI, compte tenu du nombre de décisions revenant par ailleurs au chef du Gouvernement. Cela aurait permis de ne pas remettre en cause la légitimité de l'Agence en la matière, dont l'indépendance, à terme, pourrait être envisagée. En outre, les modalités de contrôle de l'application des normes élaborées par l'ANSSI ne sont pas satisfaisantes. Nous considérons que l'Agence, qui soutient déjà considérablement les opérateurs d'importance vitale, est suffisamment dimensionnée pour effectuer les contrôles nécessaires auprès des opérateurs de services essentiels publics, sans que la charge de ces contrôles incombe à ces derniers. Les derniers points de tension résidaient dans la seconde directive relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Cette directive s'inscrit dans la continuité de la déclaration de Paris et des dispositions de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte Le régime de l'enregistrement des armes de la catégorie dite « D1 », vidé de sens, fusionne avec celui de la déclaration. La livraison d'armes est mieux encadrée, de même que la profession d'armurier, grâce aux amendements déposés en première lecture par notre rapporteur.

je me réjouis que notre assemblée ait fait un pas, ce qui nous permettra, à terme, de ratifier le protocole des Nations unies sur les armes à feu. Enfin, si nous étions tous d'accord-

Nous avons, dans notre sagesse, suivi la recommandation initiale du Conseil d'État ainsi que la rédaction de l'Assemblée nationale, en rétablissant la compétence du pouvoir réglementaire pour le classement des reproductions d'armes historiques en catégories C et D, ce qui permettra aux collectionneurs passionnés de ne pas être affectés, du moins lorsque les décrets d'application instaurant la carte de collectionneur seront pris, ce dont Mme la ministre Jacqueline Gourault nous a assurés. Au-delà des réserves que j'ai exprimées sur l'ANSSI, je considère, comme l'ensemble des membres du groupe du RDSE, que ces transpositions ainsi que les travaux de la commission mixte paritaire constituent des avancées. Nous voterons donc ce texte. La

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. Ce texte, adopté par le Sénat en décembre dernier, poursuit trois objectifs. Le premier est la transposition en droit français de la directive dite « NIS », qui impose aux entreprises européennes d'améliorer leur capacité à résister aux cyberattaques. Pour ce faire seront établies des normes communes de cybersécurité, la coopération entre les différents pays de l'Union européenne étant renforcée. L'objectif est de créer un cyberenvironnement fiable au sein de l'Union européenne, en vue de soutenir le marché intérieur. Le deuxième objectif est la transposition de la directive 2017/853 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo. Il convient de le noter, ce texte a fait l'objet d'un certain consensus, soutenu par presque tous les groupes politiques, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Espérons seulement, mes chers collègues, que ce consensus ne soit pas le résultat d'un travail parlementaire de faible qualité dû au déclenchement de la procédure accélérée et donc au peu de temps dont nous avons disposé pour appréhender un projet de loi aussi dense que complexe. J'ai eu l'occasion de le dire en première lecture, la cybersécurité, la réglementation sur les armes à feu civiles et le système de positionnement par satellite Galileo recouvrent des enjeux bien différents, qui auraient mérité d'être traités séparément dans un temps propice à un travail législatif approfondi. La commission des lois du Sénat avait d'ailleurs soulevé un risque d'inconstitutionnalité de l'article 6 de loi relatif aux obligations s'imposant aux opérateurs de services essentiels en matière de cybersécurité, tout en estimant ne pas pouvoir aller plus loin à ce stade, faute d'informations suffisantes sur le niveau de protection susceptible d'être exigé. Il semblerait que le passage du texte à l'Assemblée nationale ait permis de lever ce doute, ce qui vient confirmer, pour ceux qui en douteraient encore, tout l'intérêt de la navette et du travail législatif, tant en commission qu'en séance Finalement, seuls deux points restaient en discussion : d'une part, la directive Armes à feu, à propos de laquelle les deux chambres avaient des positions divergentes en ce qui concerne les collectionneurs d'armes historiques, et, d'autre part, la création, souhaitée par l'Assemblée nationale, d'une infraction de tentative d'acquisition ou de cession illégale d'armes, afin de permettre à la France de se mettre en conformité avec le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu. La question du contrôle des acquisitions et de la détention d'armes, tout à fait capitale à nos yeux, aurait probablement mérité un texte plus ambitieux. La directive transposée apporte certes des précisions nécessaires sur les armureries et sur la vente par correspondance, mais elle ne traite que des personnes s'inscrivant dans un cadre légal et ne s'attaque pas du tout à la problématique du trafic. Rappelons-le, ce texte a été demandé par la France après les attentats de 2015, dans le cadre de la lutte globale contre le terrorisme. Si les dispositions du texte qui nous est présenté aujourd'hui vont dans le bon sens, elles ne suffiront pas pour mener une lutte efficace contre le trafic d'armes sur notre continent. Nous devrons, exécutif et parlementaires, reprendre le travail de persuasion contre les lobbies « proarmes » avec, pour seul objectif, notre sécurité collective. C'est donc, comme en première lecture, avec un sentiment d'inachevé, que le groupe communiste républicain citoyen et écologiste soutiendra ce texte de mise en cohérence du droit interne avec les objectifs européens. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,

Concernant Galileo, le service public réglementé de radionavigation par satellite, et même si rien n'a évolué en commission mixte paritaire, c'est une réelle satisfaction de voir l'Union européenne s'émanciper progressivement du système GPS américain. L'ambition est belle, nous devions l'encourager. Pour ce qui est de la directive NIS relative à la cybersécurité, nous avons su respecter, je l'espère, l'essence de la directive, en évitant à la fois la surtransposition et la sous-transposition. Éviter ces deux écueils était essentiel, cette directive constituant la première pierre de la construction d'une stratégie globale de l'Union européenne en matière de cybersécurité. Nous ne pouvions ignorer cette première tentative d'harmonisation des législations, qui est aussi la première initiative législative de l'Union en ce domaine. Nous avions le Nous avions le devoir de ne pas rester démunis face aux menaces inhérentes à notre temps. Je vous épargnerai la longue énumération des récentes attaques ayant ébranlé des entreprises, qu'elles soient d'envergure mondiale ou plus modeste, tout en soulignant la nécessité de nous en protéger. Avec l'accélération des avancées technologiques et la connectivité croissante des objets du quotidien, il est aujourd'hui primordial de se doter de lois permettant une lutte efficace contre les cybercriminels et la fuite des données personnelles. Or cette bataille, éminemment importante, ne peut, en l'état actuel des choses, se mener et se gagner au niveau national. La puissance publique devait réagir, c'est à présent chose faite.

Grâce à ce texte, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information jouera enfin pleinement le rôle qui est le sien. Toutefois, vous vous en souvenez certainement, mes chers collègues, lors de l'examen du texte en séance publique, nous avions émis des réserves relatives à une éventuelle inconstitutionnalité de son article 6, 6, qui imposait diverses règles minimales en matière de protection des réseaux et systèmes d'information aux opérateurs de services essentiels en matière de cybersécurité. L'Assemblée nationale a évité cet écueil, en précisant juridiquement cet article, ce dont nous nous réjouissons. Concernant les dispositions sur les armes, la réunion de la commission mixte paritaire a permis de trancher deux points restant en discussion. Il y avait, d'une part, les craintes, légitimes, de voir les collectionneurs privés de leur passion et de leurs droits par la directive Armes à feu et, d'autre part, la création, par l'Assemblée nationale, d'une infraction de tentative d'acquisition ou de cession illégale d'armes. Je reviendrai sur ces deux points. Au sujet de la détention d'armes par les collectionneurs ou les sportifs, nous avions émis quelques réserves. L'objectif annoncé de la directive étant la lutte contre le trafic illicite d'armes à feu, en réaction notamment aux tragiques et récents événements terroristes qui ont ébranlé plusieurs pays de l'Union européenne, il était impensable pour nous de voir des collectionneurs privés de leur loisir par la faute d'une législation mal conçue. La commission mixte paritaire a donc tranché, et les armes historiques au sens strict du terme resteront bien dans la catégorie D. Les collectionneurs pourront donc continuer à vivre pleinement leur passion, sans risquer quelques confusions désobligeantes. Les reproductions des armes historiques, améliorées par les techniques contemporaines, et les armes neutralisées feront quant à elles l'objet d'un décret en Conseil d'État. Cette solution nous convenant autant qu'aux collectionneurs,

Enfin, le dernier sujet concernait la création, par l'Assemblée nationale, d'une infraction de tentative d'acquisition ou de cession illégale d'armes, punie des mêmes peines que l'acquisition illégale d'armes de catégorie C. Ce point précis du texte permet à la France de tenir ses engagements internationaux et de signer le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu. il semble important d'inscrire cette lutte, au même titre que celle contre la cybercriminalité, au niveau mondial. C'est tout le sens de la création de cette infraction, qui permettra, à n'en pas douter, une lutte plus efficace contre la délinquance armée et le terrorisme, tout en préservant les collectionneurs et les sportifs. Un juste équilibre a été trouvé par la commission mixte paritaire, ce dont le groupe Union centriste se réjouit. Nous pouvons désormais nous concentrer sur les textes à venir, notamment sur la question essentielle de la protection des données personnelles que j'évoquais tout à l'heure, avec le projet de loi du Gouvernement adopté hier par l'Assemblée nationale et qui sera examiné prochainement par la Haute Assemblée. Je souhaite que les débats soient aussi ouverts et constructifs qu'ils l'ont été pour le texte qui nous réunit aujourd'hui. La parole

il a fallu faire la part de ce qui relevait- c'était l'objet principal de la directive -de la protection de ce qu'on appelle les services essentiels, les activités de marché présentant une importance particulière pour la continuité de la vie sociale et économique, et le système des infrastructures, entreprises et activités d'importance vitale, qui sont déjà régulés et encadrés

apaisé » les préoccupations et les inquiétudes des collectionneurs, en procédant à un classement législatif global des armes, sous

ayant participé pour la première fois à la réunion d'une commission mixte paritaire, je suis satisfaite que celle-ci ait abouti à un accord sur ce texte de double transposition de directives et de conséquence d'une décision du Parlement européen et du Conseil

Comme nous l'a rappelé le rapporteur, que je tiens à saluer pour avoir trouvé un accord équilibré avec nos collègues députés, deux points essentiels restaient en discussion d'une part, la directive Armes à feu, à propos de laquelle les deux assemblées avaient une position divergente concernant les collectionneurs d'armes historiques d'autre part, la création, souhaitée par l'Assemblée nationale, d'une infraction de tentative d'acquisition ou de cession illégale d'armes, afin de permettre à la France de se mettre en conformité avec le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu. Concernant l'inquiétude des collectionneurs d'armes historiques, nous leur permettons, comme ils le souhaitaient, que ces armes soient classées en catégorie D par le législateur et que les reproductions d'armes historiques et les armes neutralisées soient classées par décret en Conseil d'État, l'Assemblée nationale ayant fait un pas vers le Sénat. De plus, je me réjouis que, en marge de la discussion de ce texte, le ministère de l'intérieur ait annoncé l'adoption d'une carte de collectionneur. S'agissant de l'incrimination de tentative d'acquisition illégale d'armes, il me semble opportun que nous l'ayons acceptée, ce qui permet de mettre le droit français en conformité avec le protocole des Nations unies sur les armes à feu. Enfin, conformément aux souhaits du Sénat, l'Assemblée nationale a fait un pas en avant sur les règles minimales en matière de protection des réseaux et systèmes d'information, en renforçant les garanties constitutionnelles qui l'entourent, afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines, et en précisant la liste des domaines concernés par les mesures de sécurité qui seront imposées aux opérateurs économiques essentiels. Mes chers collègues, je suis donc une sénatrice satisfaite de la méthode adoptée, qui a permis un travail approfondi et collaboratif sur des points de droit essentiels de notre législation. Personne

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement